à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission

Depuis 2017, des progrès ont été réalisés en la matière, mais les formes de fraudes évoluent rapidement, ce qui nécessite une adaptation constante du cadre législatif. Parmi les nouvelles formes de fraude,

mon collègue Olivier Jacquin, cosigné par l’ensemble du groupe socialiste, vise à limiter les écarts de salaires et à mieux partager la richesse créée au sein des entreprises.

Pour rappel, en 1979, la rétribution des chefs d’entreprise du CAC 40 était en moyenne 40 fois supérieure au salaire minimum.

L’article 15 porte sur le report de trois ans de la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Initialement prévue pour 2027, cette suppression est désormais reportée à 2030.

Dès lors, il est légitime de s’interroger sur la pertinence de cette réforme, dans un contexte où les PME, pourtant au cœur de notre tissu économique, restent en marge d’un dispositif censé les soutenir. La suppression de la CVAE entraîne également une perte de recettes pour les collectivités locales, partiellement compensée par une fraction de TVA, ainsi qu’une perte pour l’État, alors que, manifestement, les recettes fiscales lui font cruellement défaut.

publiques locales. En 2021, sous l’impulsion du président Macron, la CVAE a été divisée par deux.

Il n’est pas membre de notre groupe ni de notre sensibilité politique. Il estimait que le report de trois ans n’avait absolument aucun sens et jugeait que cette suppression était soit un outil de relance économique

Cette volonté de proroger l’existence de la CVAE, dont le précédent gouvernement avait décidé l’extinction, constitue un très mauvais message adressé à nos entreprises. Ces impôts représentent des charges inutiles et coûteuses, peu propices à la réindustrialisation du pays, objectif central que nous défendons.

n° I 1186. Par cet amendement, nous proposons le rétablissement graduel de la CVAE pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard

locales. Afin d’assurer une stricte neutralité pour les parties prenantes, il est proposé de maintenir à due concurrence l’allocation aux collectivités d’une quote part de TVA :

lequel vise précisément à maintenir un lien entre l’installation des entreprises sur le territoire et le produit fiscal perçu. En gelant la quote part de TVA allouée aux collectivités, l’article 31 du du présent projet de loi de finances vient ôter au Fnaet de nouvelles ressources. En cela, il réduit l’intéressement des communes et de leurs groupements à l’accueil d’entreprises, en totale contradiction avec

Mes chers collègues, soutenir cet amendement, c’est faire preuve de bon sens et promouvoir une justice fiscale indispensable à la vie de nos territoires.

dernière taxe, présentée comme la recette idoine pour compenser les collectivités, est désormais gelée, à rebours des promesses qui avaient été faites par les ministres.

ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). Il s’agit d’un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 mètres carrés réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, à l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon desdits produits. N’étant pas ouverts à la circulation des clients, les ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la Tascom. Or ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non assujettissement qui n’est pas justifié, alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail. Les ainsi que la vente à distance, notamment au travers des sites de commerce en ligne, se sont très fortement développés en France.

Ainsi, les et entrepôts de l’e commerce, qui génèrent un chiffre d’affaires considérable, ne sont pas soumis à la Tascom, contrairement aux commerces physiques. Cette situation constitue une injustice – vous en conviendrez, monsieur le ministre – et entrave les efforts pour équilibrer le développement économique des territoires. Depuis 2016, le chiffre d’affaires de l’e commerce en France a doublé, atteignant près de 150 milliards d’euros en 2023. Pourtant, ces activités échappent largement à la fiscalité locale, car leur localisation logistique ou numérique réduit l’assiette taxable. Par exemple, les collectent principalement la TVA des mécanismes simplifiés, laissant les collectivités sans retombées fiscales significatives. Les, qui se sont multipliés plus de 7 000 en 2023 –, occupent des surfaces commerciales comparables aux magasins traditionnels, mais ne sont pas soumis aux mêmes charges, bien qu’ils contribuent à l’artificialisation des sols et modifient les flux économiques locaux.

au même titre que les commerces de proximité.

denses, où les opérateurs ont réalisé les installations nécessaires, et les zones moins denses, qui sont devenues des zones blanches, notamment en montagne. Pour essayer de remédier à cette situation et réduire ces écarts,

économiques. Dans un contexte de crise des finances publiques, il n’est plus acceptable d’engager des montants substantiels d’argent public à destination des entreprises sans contrepartie et sans considération pour l’intérêt général. Dans cette perspective, le dispositif retenu cible des entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière. Sont ainsi concernées les sociétés cotées de plus de 500 salariés, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 40 millions d’euros, ainsi que les sociétés non cotées de plus de 500 salariés, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros. La philosophie des auteurs du présent amendement est de suivre une logique d’ensemble en appliquant la conditionnalité à toutes les aides publiques, que ce soit les subventions, les garanties de prêt, les garanties publiques pour le commerce extérieur, l’éligibilité à tous les crédits d’impôt sur l’impôt sur les sociétés, notamment le crédit d’impôt recherche, les participations de l’Agence des participations de l’État (APE) ou celles de Bpifrance. De plus, l’accès à la commande publique, forme dérivée d’aide publique, est incorporé dans le dispositif. Le présent amendement vise donc à conditionner plus sérieusement les aides publiques en fonction de critères plus exigeants.

Jean Jacques Panunzi. Cet amendement a pour objet de soutenir l’investissement des pêcheurs insulaires confrontés au nécessaire renouvellement de leurs équipements pour rester compétitifs et assurer la transmission aux jeunes générations.

le prix de la cantine est fonction du quotient familial. Dès lors, il semble important que la taxe de séjour soit proportionnelle à la qualité du logement

par catégorie d’établissement, afin que les collectivités puissent définir des taux selon le prix de la nuitée, dans une fourchette allant de 0,5 % à 5 % du montant facturé pour tous les hébergements de tourisme. Un taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement. Cet amendement tend à maintenir la faculté de moduler le taux proportionnel en fonction de la catégorie d’hébergement afin de faire évoluer le tarif de la taxe de séjour en fonction du prestige des hébergements et pour tenir compte des spécificités locales du territoire.

Monsieur le ministre,

707 vise à rendre systématique et obligatoire l’accord préalable de l’administration fiscale sur la politique de prix de transfert menée par une entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.

Tout en étant souple et incitatif, ce dispositif leur offre un levier essentiel pour traverser les périodes difficiles. Toutefois, le secteur agricole est confronté à une intensification desdites crises. Ces épisodes Ces épisodes fragilisent de manière récurrente les exploitations et les mènent parfois jusqu’à la cessation d’activité. Afin de soutenir concrètement les exploitants, nous proposons que lorsque les sommes issues de la DEP sont utilisées pour couvrir les dépenses liées à ces risques, seuls 50 % des montants déduits soient réintégrés dans le résultat fiscal de l’exploitation. Cette mesure vise à garantir une trésorerie supplémentaire aux exploitants faisant face à ces événements imprévisibles. En adoptant cette modification, nous renforcerons l’efficacité de la DEP, assurant ainsi une aide tangible à nos agriculteurs pour mieux faire face aux crises qui menacent leur avenir, la sécurité alimentaire et la souveraineté agricole de notre pays. La

Ce seuil se surajoute inutilement à la limitation à 70 % de la réintégration des sommes. L’épargne de précaution doit pouvoir être mobilisée en cas d’aléa de très forte intensité afin de ne pas mettre en péril les exploitations de nos agriculteurs.

lait. Ce dispositif nécessite des ajustements pour être pleinement efficace. Premièrement, il est proposé de plafonner le montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas, à la clôture de l’exercice, partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles, et ce de manière dégressive.

Deuxièmement, il s’agirait de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle qui est constatée sur l’exercice de constitution de la provision.

afin de sécuriser le revenu de l’exploitant, il n’en demeure pas moins que sa mise en œuvre reste très compliquée sur le terrain pour la production de viande bovine. Pour tenir compte des difficultés que rencontrent les exploitants dans l’établissement de ces contrats, que ce soit pour la fixation des prix il est proposé de renvoyer à un décret les conditions de la contractualisation, en prévoyant notamment une progression dans le taux de contractualisation par l’éleveur de sa production de viande.

à l’accroissement du cheptel au sein de systèmes d’élevage herbagers. Il s’agit d’encourager des pratiques agricoles durables qui préservent l’environnement, favorisent la biodiversité et sont plus respectueuses du bien être animal.

à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socioéconomiques. Ainsi, le dispositif de cet amendement, adopté par l’Assemblée nationale sur l’initiative du groupe Les Démocrates, avant que la première partie du projet

Cet amendement vise à instaurer un système de bonus malus sur les produits alimentaires en fonction de la transparence des informations affichées sur leur emballage. Ce système repose sur trois critères essentiels : la qualité nutritionnelle, l’impact environnemental et l’origine des matières premières et du lieu de transformation.

dans nos supermarchés et de réduire le coût social, écologique et budgétaire des produits alimentaires de mauvaise qualité environnementale et nutritionnelle. Il est ainsi proposé d’instaurer une taxe de 10 centimes

En France, 70 % du couvert forestier est privé. Nous ne pouvons pas faire l’impasse sur les enjeux de la préservation de la biodiversité dans les forêts privées dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité

un rôle crucial dans les territoires ruraux forestiers, notamment en Nouvelle Aquitaine. Il s’agit donc de relever les plafonds proposés de 6 250 euros à 15 000 euros pour une personne seule, et de 12 500 euros à 30 000 euros pour un couple.

Michaël Weber. L’exploitation massive des grumes vers l’Asie est un phénomène largement connu et dénoncé sur toutes les travées de cet hémicycle. Chaque année, des milliers de tonnes de bois produit en France sont exportées essentiellement vers la Chine. Ce bois y est transformé et retourne en Europe sous la forme de produits manufacturés. Cette incongruité de l’économie mondialisée affecte fortement l’emploi et fragilise l’approvisionnement des scieries en France, sans parler de son bilan carbone catastrophique. Pour remédier à cette situation, cet amendement vise à conditionner les aides publiques à l’engagement de vendre les coupes sur le territoire de l’Union européenne pour inciter à la transformation du bois en France ou en Europe. C’est ainsi que l’argent public cessera enfin de financer l’hémorragie du bois français !

plus durable. Dans sa forme actuelle, le Defi « travaux » n’offre aucune incitation supplémentaire aux pratiques favorables à la biodiversité et à la protection des sols, telle que la sylviculture mélangée à couvert continu. Nous proposons donc d’ajouter un bonus permettant de bénéficier d’un crédit d’impôt de 40 % au lieu de 25 % pour la réalisation de travaux de sylviculture mélangée à couvert continu

forestiers, qu’ils soient engagés dans une gestion durable de leur bien ou non. Cet amendement vise à offrir une incitation supplémentaire pour les propriétaires qui s’engagent à gérer durablement leur forêt en maintenant un couvert forestier continu, en portant ce crédit d’impôt à 40 %.